Aucune disposition n'est prévue pour prendre en compte les nuisances quotidiennes subies par les riverains de voies ferroviaires, de jour et de nuit, lors des passages des trains à plus de 250 kilomètres J'ai une pensée particulière pour les riverains girondins du TGV Bordeaux-Paris. Pourtant, aux contraintes sonores traditionnelles, s'ajoutent bien des contraintes vibratoires, qui présentent de nombreux désagréments tant dans la gêne ressentie par les habitants que dans la fragilisation des structures des bâtiments et des équipements sensibles. Faute de normes applicables en la matière, SNCF Réseau est contraint de s'inspirer d'autres dispositions, notamment de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, pour déterminer les dommages provoqués sur les biens. Malheureusement, pour déterminer les gênes perçues par les personnes, le coût humain et social, la norme ISO 2631 ne fixe aucune valeur seuil. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'Anses, le reconnaît volontiers elle-même : peu de données existent sur les vibrations engendrées par les infrastructures de transport. Cet amendement vise donc à ce que les nuisances provoquées par les vibrations aux abords des infrastructures de transport ferroviaire fassent l'objet d'un rapport du Gouvernement remis au Parlement. L'objectif est de pouvoir disposer de bases scientifiques solides, avant d'envisager toute évolution réglementaire en la matière. Pour autant, il faut que les nuisances vibratoires soient à l'avenir prises en compte dans la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et qu'une unité de mesure spécifique

L'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires fixe deux plages horaires de référence, diurne et nocturne, sur lesquelles est mesurée une moyenne du niveau continu de pression acoustique en décibels. Le premier écueil de ce système de mesure est qu'il ne prend pas en compte les « pics de bruit » correspondant aux passages de train à près de 300 kilomètres par heure. C'est pourquoi je me réjouis de l'adoption de mon amendement en commission visant à prendre en compte ces indicateurs événementiels qui, comme le reconnaît le rapport gouvernemental du 27 juin dernier, ont des effets néfastes à long terme sur les riverains exposés. Le deuxième écueil auquel cet amendement s'attaque est l'instauration en 1999, soit il y a vingt ans, d'un système de mesure des contraintes sonores en décibels. L'échelle des décibels est non pas linéaire, mais logarithmique. Cela veut dire que la valeur du bruit mesuré lors du passage de deux trains à un endroit donné équivaut non pas à la somme des valeurs mesurées, mais à la valeur corrigée d'un premier bruit. Par conséquent, la somme du bruit de deux trains avec chacun une pression acoustique à 60 décibels donnera un bruit cumulé mesuré à 63 décibels. Par exemple, si une habitation est située entre une ligne à grande vitesse et une autoroute- je pense une fois encore à des villes situées à proximité de Bordeaux -, la source la plus bruyante sera prise en compte dans l'évaluation de la nuisance sonore subie par le foyer. Si l'autoroute prend le dessus, c'est comme si la ligne à grande vitesse n'existait pas ! Afin de pallier cette incohérence, le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport relatif à l'amélioration de la mesure et de l'évaluation des nuisances sonores cumulées provoquées par les transports ferroviaires. L'objectif est, encore une fois, de pouvoir disposer de bases scientifiques solides avant d'envisager toute évolution réglementaire en la matière pour que les mesures des nuisances sonores aux alentours des chemins de fer puissent retranscrire la véritable

complexes. Notre politique en termes de nuisances sonores autour des infrastructures de transport se déploie sur trois niveaux : le bruit émis par les nouvelles infrastructures prises individuellement est strictement limité par la réglementation ; les constructions nouvelles doivent tenir compte des infrastructures à proximité ; les situations de points noirs créées avant la mise en oeuvre des réglementations en la matière sont progressivement traitées. Dans le domaine du ferroviaire, comme vous l'avez rappelé et comme cela a été évoqué à l'occasion d'autres amendements, la réglementation se base sur un bruit moyen, sans prendre en compte les pics d'émission. Le Gouvernement est parfaitement conscient des difficultés que cela peut engendrer

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Ademe, a remis en décembre 2016 un rapport au Parlement, disponible en ligne, sur l'évaluation de l'impact environnemental du transport par autocar.

autocars ont un impact sur ce bilan environnemental. Cet amendement vise à prévoir qu'un nouveau rapport soit remis par l'Ademe au Parlement sur l'impact environnemental du secteur. Il se pérenniserait ensuite sous la forme d'un rapport triennal.

d'habilitation concerne l'adaptation de notre droit à la réglementation européenne en matière de contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur. Je regrette que Je regrette que les textes des ordonnances n'aient pas pu nous être transmis en amont de l'examen du texte, d'autant que les règlements de 2013 sont applicables depuis 2016 et que le règlement de 2018 le sera au 1 septembre 2020. 1 septembre 2020. Néanmoins, des indications assez précises m'ont été transmises concernant le fonctionnement du futur service à compétence nationale qui sera créé- le service de surveillance du marché des véhicules -et qui sera chargé de contrôles réguliers. Toutes ces précisions figurent dans le rapport de la commission. Il y a urgence à adapter notre droit : avis défavorable.

telle mesure. Je pense notamment à l'Angleterre, où très clairement le prix des pièces n'a pas chuté. Les marges des réparateurs indépendants qui ne sont pas dans les réseaux de concessionnaires ont augmenté, mais les prix pour le public n'ont pas baissé. L'économie réalisée

Le Premier ministre a annoncé le 5 mars dernier qu'il voulait une évolution des règles encadrant les conditions dans lesquelles les équipementiers peuvent fabriquer des pièces de rechange dites « équivalentes aux pièces de marque constructeur. Ces mesures prendraient le relais d'une première initiative que les constructeurs et les équipementiers de première monte ont prise en 2017 en signant une charte

conforterait davantage les équipementiers. Dernier argument : les dessins et modèles sont une question de propriété industrielle et commerciale, ce qu'on appelle en droit de la propriété « l'unité de l'art

résultat de décennies de sous-investissements, nécessitait un sévère rattrapage. Faisant siennes les conclusions d'un audit externe réalisé sur les besoins de restauration de l'infrastructure fluviale, le COI a indiqué que, pour maintenir la fonction navigation sur l'essentiel du réseau, un budget de 245 millions d'euros par an serait nécessaire pendant dix ans. Ce chiffre n'inclut pas le budget de 30 millions d'euros prévu par VNF pour la modernisation du réseau. Le Conseil d'orientation des infrastructures a évalué qu'un scénario minimaliste réduit à 201 millions et 30 millions d'euros d'autofinancement pour la régénération, impliquerait d'abandonner la fonction navigation sur 20 % du réseau.

en 2027 avec les fonds propres et les cofinancements supposés. Mais ces montants incluent les 30 millions d'euros par an prévus pour la modernisation. Ainsi, en 2027, 160 millions au mieux, consacrés à la régénération du réseau, au lieu des 245 millions d'euros par an nécessaires. Ce scénario signifie qu'une part importante du réseau devra être fermée à la navigation, privant de nombreux territoires d'une desserte fluviale pour le transport comme pour le tourisme. À l'heure où l'on enregistre un dérèglement climatique qui dépasse tous les pronostics, il est nécessaire de conserver l'intégralité d'un réseau qui permet d'assurer des prestations de transport trois à quatre fois moins émettrices de gaz à effet de serre que le transport routier. Le nouveau scénario propose de viser à l'horizon de 2023 un budget de 245 millions pour la régénération, auquel s'ajouteraient 30 millions d'euros pour la modernisation, soit 275 millions d'euros Cet amendement tend à rétablir un titre que nous avons déplacé à l'article 1 A. Nous avons déjà eu le débat sur le fond des crédits dédiés au maritime et au fluvial sur des amendements similaires au titre I A. Je rappelle que le budget de l'Afitf concernant le fluvial est passé de 50 millions à 80 millions d'euros,

est le sens des audits que j'ai demandés, dès ma prise de fonctions, sur les réseaux ferroviaire, fluvial et routier. Ces audits font tous apparaître que nous avons pris, pendant des décennies, un retard important en termes d'entretien et de régénération de nos réseaux-

est à M. Rémi Féraud. À l'instar de l'amendement que j'avais présenté à l'article 28, celui-ci vise à rendre les plus opérants possible le contrôle et la verbalisation des éventuelles infractions dans les zones à faibles émissions, les zones à trafic limité et les aires piétonnes lorsque les véhicules qui ne sont pas autorisés les empruntent. L'objet de cet amendement est de mettre en place la vidéoverbalisation de ces infractions. À cet vise à permettre aux services de police et de gendarmerie, aux services de police municipale et, à Paris, au service dont relèvent actuellement les agents de surveillance de Paris de consulter le fichier des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées et, si c'est nécessaire,

prévoit, à l'article 16, des dispositions spécifiques pour les zones à faibles émissions. En conséquence, un décret en Conseil d'État sera pris pour compléter la liste des infractions constatables par la vidéoprotection. Enfin, les forces de l'ordre disposent déjà d'un droit d'accès au système d'immatriculation des véhicules.

Après bientôt trois ans d'effectivité, la loi Macron a montré une limite en matière d'apprentissage de la conduite dématérialisée, avec l'apparition des acteurs en ligne. En effet, ces plateformes n'ont pas de local et font souvent appel à des formateurs sous statut d'auto-entrepreneur. Cette concurrence donne lieu à un important contentieux entre ces deux types de structure et n'améliore pas la situation. Outre la question de l'agrément préfectoral, qui fait l'objet de l'amendement que je vous présenterai dans quelques instants, il est ici question du statut de salarié. salarié. Ces personnes disposent en effet d'un statut fiscal contournant le paiement des charges sociales et qui peut répondre à une définition du travail dissimulé, un peu à l'instar des employés du BTP qui ont ce statut le week-end, par exemple, et qui disposent des moyens de leur entreprise sans en avoir les charges. J'avais d'ailleurs déposé un amendement sur ce sujet en commission spéciale lors de l'examen Par ailleurs, les enjeux en termes de sécurité et d'assurance sont revus à la baisse, avec une prise en charge des élèves et des prix extrêmement variables en fonction de la structure choisie. Des dépôts de plaintes ont été enregistrés, notamment dans les Alpes-Maritimes, sur le travail dissimulé à l'encontre de l'un des leaders en ligne, Ornikar. Enfin, la situation professionnelle des moniteurs est à souligner, puisque le traitement, la rémunération et la protection sociale sont très différents en fonction de leur statut de salarié ou d'auto-entrepreneur, ce qui aboutit de fait à une rupture d'égalité et à une concurrence déloyale. C'est un vrai sujet, qui a des conséquences importantes sur la concurrence dans ce secteur, ainsi qu'en matière de rémunération et de protection sociale pour les professionnels concernés. Un travail est en cours pour définir au niveau législatif de nouveaux principes en matière de sécurité routière et d'enseignement de la conduite.

est l'avis du Gouvernement ? Il n'est pas possible, au regard des traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'interdire purement et simplement l'activité des auto-entrepreneurs dans le domaine de l'éducation routière. Par ailleurs, des décisions judiciaires sont attendues, qui permettront de préciser dans quelle mesure le statut d'auto-entrepreneur pour les moniteurs est susceptible d'être, ou non, requalifié, ainsi que les conséquences qu'il faudrait en tirer en termes de répartition des responsabilités entre les deux parties. Dans l'attente de ces décisions, il ne paraît pas opportun de légiférer sur ce sujet. De façon plus générale, cela a été rappelé, une mission a été confiée à la députée Françoise Dumas, qui a remis un rapport au Premier ministre le 12 février 2019. Nous avons engagé une concertation avec les organisations professionnelles du secteur de l'éducation routière,

est à Mme la ministre. Cet amendement vise à permettre aux forces de l'ordre, sur autorisation du préfet, de procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière d'un véhicule pendant une durée de sept jours, pour écarter provisoirement de la route l'auteur d'un délit de conduite sous l'influence de l'alcool, de conduite après usage de stupéfiants ou de conduite sans permis de conduire.

zones rurales. Il sera toujours possible de faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière judiciaires du véhicule, dans le cadre d'une procédure faisant intervenir le procureur de la République. L'avis est donc défavorable. La parole

sur une position qui était celle de la commission des lois et de la commission du développement durable. Vous proposez de substituer à l'autorité judiciaire, c'est-à-dire le procureur qui peut à tout moment prendre cette décision,

et que l'on ne saurait remplacer d'une manière courante la mesure exceptionnelle, créée en 2011, qu'est le recours à une autorisation administrative du préfet. nous donne donc les moyens de sanctionner, comme vous souhaitez le faire, en utilisant l'autorité judiciaire et non l'autorité administrative. À titre personnel, je voterai donc contre cet amendement. La parole est

Les entreprises de transport souhaitent pouvoir disposer de caméras frontales embarquées à l'avant de leur matériel roulant, afin de pouvoir filmer, à la fois, la circulation et la voirie. En

embarquées, notamment à l'avant des tramways et des bus, qui visualisent la voie publique, pour améliorer la qualité du service public délivré et offrir de meilleures garanties en termes de sécurité routière. La présence de ces caméras La présence de ces caméras permettrait en effet de comprendre les causes d'un incident technique ou d'un accident impliquant des éléments extérieurs- piétons, voitures ... -et, dès lors, de prendre des mesures destinées à prévenir ce type d'incident ou d'accident, pour se conformer, notamment, aux préconisations du Bureau

pas moins quelques interrogations. D'abord, il est prévu non seulement un enregistrement, mais également une transmission d'images de la voie publique. S'agit-il d'une transmission en direct ?

essentielle. Enfin, il serait possible de conserver sans limitation de durée les enregistrements effectués, sous réserve de leur anonymisation. Outre la difficulté technique que nous connaissons pour procéder à cette anonymisation- nous en avons débattu au sujet des articles précédents -, je m'interroge sur la justification de cette conservation durable d'enregistrements de la voie publique, qui n'est prévue dans aucun système d'enregistrement vidéo. du Gouvernement ? Je vois que notre grand opérateur de transport veut se donner les moyens de régler les incidents qui peuvent survenir- je sais qu'ils sont nombreux -, mais je pense qu'il n'a pas suffisamment pris en compte les atteintes aux libertés individuelles que ces dispositions pourraient engendrer. Ces sujets sont extrêmement sensibles. L'utilisation de caméras de vidéoprotection est strictement encadrée

de l'utilisation de caméras mobiles, ce qui a conduit à prévoir un cadre très strict, notamment pour l'utilisation par les forces de l'ordre de caméras-piétons, mais aussi pour l'expérimentation de ces outils par d'autres acteurs. En de caméras sur les véhicules de transport en commun qui filmeraient l'ensemble de la chaussée et de ses abords ne paraît pas nécessaire ni proportionné à l'objectif assigné à ces dispositifs ; il constituerait une atteinte trop importante aux libertés individuelles, même dans le cadre d'une expérimentation. Je vous suggère donc de retirer ces amendements,

ou non. Or, si la perte totale de points occasionne pour tous le retrait du permis, pour les conducteurs routiers, elle entraîne également la perte de leur emploi. Cette situation est d'autant plus problématique que le secteur du transport fait face à une pénurie de chauffeurs. si la France compte 345 000 chauffeurs routiers, plus de 16 000 postes sont aujourd'hui à pourvoir. Aussi proposons-nous des modalités spécifiques de récupération de points pour les conducteurs professionnels des transports routiers, afin de leur permettre de conserver leur emploi.

serait en réalité un droit de transgression pour certaines catégories de personnes sur la route, d'autant que la majorité des professionnels sont respectueux des règles. Cette différence de traitement ne se justifie pas au regard de la nécessité d'assurer la sécurité routière.

qui est de permettre l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles, non de corriger les conséquences d'infractions routières. Quant à la formation continue, c'est un sujet dont nous discutons avec les organisations de transport routier. La réflexion n'est pas aboutie au niveau interministériel, notamment sur les règles qu'il faudrait fixer dans le cadre des formations continues obligatoires pour qu'elles répondent aux mêmes exigences que les

vote. Au risque de rompre la belle unanimité d'il y a quelques instants, je suis plutôt contre ces amendements. Il est bien évident qu'il y a une problématique : celle des chauffeurs routiers,

entre les auto-écoles dites classiques, disposant d'un local, et celles qui opèrent exclusivement en ligne. Si un rapport d'information de l'Assemblée nationale consacré au suivi de la loi dite Macron propose de rappeler dans la partie législative du code de la route que l'agrément délivré aux professionnels par le préfet est d'ordre national, il semble plus cohérent de laisser au Conseil d'État le soin de définir l'agrément, afin de donner aux préfets la possibilité d'arbitrer les demandes d'agrément entre des acteurs qui ne disposent pas des mêmes moyens

au détriment des élèves comme des conditions de travail des professionnels. La disparition des auto-écoles traditionnelles au profit de nouveaux acteurs en ligne n'est en rien une garantie d'efficacité pour les élèves. Elle risque, à terme, de réduire la qualité de la formation dans les territoires. La partie réglementaire du code de la route déterminant que l'agrément du préfet a une portée nationale, compte tenu de la nature de la route, il paraît cohérent de laisser le Conseil d'État définir cet agrément et d'en fixer les limites, afin de laisser les acteurs se développer à leur juste place en fonction de leur stratégie commerciale et professionnelle, plutôt que d'imposer un des deux modèles sans concertation. La délivrance d'un agrément doit protéger l'élève en lui garantissant que l'exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires localement pour lui dispenser des formations répondant aux exigences assurantielles.,

dans un département en particulier ? Quels contrôles administratifs mener dans ce cas ? Le Conseil d'État mettrait ainsi fin au conflit.

L'exploitation d'une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d'un agrément préfectoral qui protège l'élève en lui garantissant que l'exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires pour dispenser des formations répondant aux exigences réglementaires. Afin d'obtenir l'agrément préfectoral, l'établissement doit justifier du respect d'un certain nombre d'exigences, garantes de la bonne qualité de l'information dispensée. En particulier, il doit disposer d'un local permettant des enseignements théoriques et un ancrage territorial. Parce qu'elles délivrent l'agrément et disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à même d'assurer le respect de ces obligations légales. Il convient donc de s'assurer que la loi précise bien que l'agrément délivré est de portée départementale, en clarifiant l'article L. 213-1 du code de la route. autre solution rendrait toute volonté de contrôle inopérante et nierait l'intérêt pédagogique du local. Cette proximité et cette capacité de contrôle conditionnent une haute qualité d'éducation routière et garantissent ainsi un haut niveau de sécurité routière.

Notre amendement visait à mener une expérimentation en matière de covoiturage entre autorités organisatrices de la mobilité et auto-écoles, aux fins d'intégrer l'apprentissage du covoiturage au sein de l'ensemble des programmes d'éducation et de formation en matière de sécurité routière. L'idée étant que, à terme, l'apprentissage du covoiturage soit intégré au sein du dernier module du REMC. Par ailleurs, cet amendement tendait à permettre, simultanément à l'apprentissage du covoiturage, le transport de tiers, afin d'encourager une pratique innovante à petite échelle de répondre de manière pragmatique aux problèmes de mobilité des territoires peu denses, qui ne disposent pas ou peu de transports collectifs et sur lesquels le covoiturage en tant que tel peut être difficile à développer efficacement. Je sais que vous explorez en ce moment des pistes innovantes de mobilité dans les territoires ruraux et périurbains, dans le cadre du projet. La solution que nous proposions s'intégrait exactement dans l'approche de rural à l'égard de laquelle j'ai compris votre bienveillance.

loyales. L'agrément pour les auto-écoles sous forme de plateformes en ligne pose effectivement des questions, dans la mesure où le principe, aujourd'hui, est que les agréments sont délivrés par le préfet du département, mais ont une portée nationale.

l'engagement de revenir devant le Parlement pour prévoir des dispositions permettant de gérer dans les meilleures conditions possible les agréments des auto-écoles en ligne.

L'article 2 de la loi Le Roux-Savary du 22 mars 2016 a autorisé à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1 janvier 2017, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

2018, 3 367 missions avaient déjà été menées avec l'appui de ces caméras-piétons. Environ 10 % de ces missions ont fait l'objet d'un déclenchement du dispositif. Les caméras permettent d'apaiser les tensions et de sécuriser les missions des agents, en limitant les risques de comportements agressifs. Elles apportent également la preuve du bien-fondé d'une intervention et contribuent à améliorer la sécurité des usagers.

L'expérimentation de la SNCF prendra fin le 1 janvier 2020. D'ici là, il convient de ne pas poursuivre une expérimentation devenue inutile et de pérenniser le dispositif pour sécuriser les transports, parce que tout cela fonctionne très bien. Quel est l'avis de la commission ?

comme le prévoit l'article 10 du décret du 23 septembre 2016. De plus, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a demandé, dans sa délibération du 8 décembre 2016 relative au projet de décret précité, à être consultée préalablement à la pérennisation du dispositif.

mis en place pour les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. La loi Savary a permis l'usage de caméras-piétons à titre expérimental pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2019. Entre la prise de connaissances du

: La parole est à M. Alain Fouché. Cet amendement vise à permettre à l'ensemble des contrôleurs et vérificateurs de titres des entreprises de transport de voyageurs d'utiliser des caméras individuelles portatives dans l'exercice de leurs missions, afin de faire progresser la sûreté sur les réseaux de transport de voyageurs. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP expérimentent l'utilisation de caméras mobiles depuis le mois de février 2018. Les résultats sont très concluants. La présence des caméras permet en effet d'apaiser les tensions et de sécuriser les missions des agents. Le bénéfice de ce dispositif en termes de sécurité publique est connu et reconnu ; une expérimentation est donc inutile. L'objet du présent amendement est d'étendre l'utilisation des caméras-piétons à l'ensemble des agents assermentés des exploitants du service de transport. En effet, ces entreprises sont aujourd'hui tentées de recourir

La loi de 2016, que nous avons évoquée, dite loi Savary, précise dans l'article L. 2251-4-1 du code des transports que seuls les agents de la SUGE et du GPSR sont autorisés à utiliser des caméras-piétons, excluant ainsi tout agent de contrôle assermenté, alors que beaucoup de territoires souhaitent équiper leurs agents de contrôle assermentés. Malgré tout, certains responsables de réseaux de transport passent outre, avec l'accord du représentant de l'État dans le département- il faut quand même le préciser -, tandis que d'autres reçoivent un avis négatif. Depuis leur déploiement, les caméras-piétons ont prouvé leur efficacité dans la lutte pour la réduction des agressions physiques et verbales que subissent les agents lors du contrôle de contrevenants. Les collectivités ayant pu équiper leurs agents ont vu baisser drastiquement le nombre d'agressions et incivilités envers ces derniers. Cet outil permet d'apaiser les tensions lors du contrôle dès lors que l'agent prévient l'usager,

Sous le couvert d'une convention entre le responsable du réseau de transport public et la préfecture, la sécurité publique du Rhône visionne en direct les images de toutes leurs caméras. la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016, dite loi Savary, que l'on a évoquée, l'article L. 1632-2-1 du code des transports dispose que « la transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport ». Compte tenu du risque terroriste, il est nécessaire de revoir les modalités de déport permanent des images en temps réel du réseau de transport public aux forces de l'ordre- police, gendarmerie et police municipale -pour assouplir les cas dans lesquels ce déport est assuré. Un conventionnement tripartite entre les réseaux de transport, les forces de l'ordre et l'État permettra d'encadrer ces modalités. Compte tenu du risque

? Cet amendement vise à procéder à une extension importante des possibilités de transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs, en supprimant le critère de la gravité de l'incident en cause. Au regard Au regard des arguments que vous venez de développer sur le terrorisme, j'indique que la notion de gravité est aujourd'hui mentionnée. Il s'agit d'informations sensibles pour les citoyens, auxquelles les forces de l'ordre pourraient avoir accès en temps réel. ce dispositif ne me semble pas proportionné à l'atteinte résultant pour la vie privée. En conséquence, l'avis est défavorable.

ne vise que les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d'une entreprise de transport public de personnes ou d'une entreprise de transport de marchandises dangereuses, à l'exclusion du gestionnaire d'infrastructure ou du groupe public ferroviaire. ce texte retient le vocable d'« emplois », sans préciser si ces derniers concernent exclusivement les salariés des entreprises concernées. Ainsi, cet article doit être modifié afin, d'une part, de viser le gestionnaire d'infrastructure ou du groupe public ferroviaire et, d'autre part, de préciser quelles personnes peuvent faire l'objet d'une telle enquête administrative, en y incluant incluant les salariés des entreprises visées ou du gestionnaire d'infrastructure, mais également les personnels mis à disposition ainsi que les personnels des sous-traitants qui interviennent au sein des entreprises citées.

Ces amendements prévoient d'élargir sensiblement le champ de l'article visé du code de la sécurité intérieure, qui couvre déjà de très nombreux cas. En 2018, le service national des enquêtes administratives de sécurité avait fait état de 8 473 demandes, dont 72 % ont été émises dans un contexte de recrutement et 28 % formulées à l'occasion d'un changement d'affectation interne. C'est déjà un volume très important, mais la sécurité est sans doute à ce prix. Si ces amendements étaient adoptés, il en résulterait une charge si importante pour le ministère de l'intérieur que ce dispositif serait particulièrement difficile à appliquer, non seulement par le ministère, mais également par les opérateurs concernés, qui auraient beaucoup de mal à consulter en temps réel pour les sous-traitants et les exploitants,

: La parole est à M. Alain Fouché. La loi Le Roux-Savary du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. L'enquête est réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité après consultation de plusieurs fichiers d'État. Les avis d'incompatibilité sont rendus à l'encontre des personnes dont le comportement fait craindre à l'État à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, d'un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Cet avis d'incompatibilité peut faire l'objet d'un recours administratif. Dans une telle situation, l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure prévoit l'obligation pour l'employeur de reclasser l'agent- c'est très dangereux ! -dans un autre emploi. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié que l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.

Il apparaît totalement inopportun de reclasser dans l'entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que le comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. de celle-ci dans une autre fonction, quand bien même cette dernière ne serait pas considérée comme sensible, fait tout de même courir des risques pour la sécurité des personnes transportées et celle de ses collègues. La seule détention d'une carte professionnelle SNCF par un agent identifié comme dangereux est problématique, puisqu'il aura accès à tous les services. En conséquence, le licenciement d'un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l'entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement. C'est d'ailleurs le cas pour certains emplois

difficiles dans les grandes entreprises publiques de transport et ces dernières souhaitent effectivement se séparer des personnes désignées par les autorités publiques comme dangereuses.

en termes de rédaction : il y a une répétition au septième alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, ce qui introduit une confusion quant à la suppression de l'obligation de reclassement.

peuvent faire l'objet de mesures d'éviction, à condition qu'il y ait préalablement une solution en termes d'hébergement. Par ailleurs, je sais que la présidente d'Île-de-France Mobilités

M. Michel Vaspart. Mon amendement est complémentaire de celui de M. Karoutchi. Lorsque le résultat d'une enquête fait apparaître que le comportement d'un salarié est incompatible avec l'exercice de ses missions, et en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus du salarié, l'employeur est tenu d'engager une procédure de licenciement. Le motif du licenciement n'étant pas disciplinaire, l'employeur doit assumer le coût financier et le risque de contentieux liés à la procédure de licenciement. Cet amendement tend à ce que la rupture du contrat de travail consécutive à une enquête administrative effectuée par le ministère de l'intérieur n'entre pas dans le cadre légal du licenciement. L'entreprise n'a pas à supporter le coût de la décision administrative ni les risques de contentieux afférents, alors qu'elle n'y est strictement pour rien.

et de veiller au bon fonctionnement du service. Dans la perspective de l'ouverture à la concurrence, l'article 33 vise à adapter le périmètre d'intervention des services de sécurité de la RATP et à encadrer les conditions d'exercice de cette mission pour qu'elles soient transparentes, équitables et non discriminatoires. Ladite mission doit notamment être séparée sur le plan comptable des activités d'exploitant de service de transport public de voyageurs et de gestionnaire d'infrastructure dévolues à la RATP. Nous considérons qu'il n'est pas nécessaire

le GPSR soit séparé de l'établissement public industriel et commercial RATP pour remplir ses missions, y compris postérieurement à l'ouverture à la concurrence. L'article 33 prévoit une séparation comptable exigences en termes de concurrence et de transparence de l'information. Toutefois, la précision que vous proposez reviendrait à s'immiscer dans la gestion du groupe RATP, alors que ce dernier pourrait choisir de filialiser cette activité si cela lui paraît nécessaire à un moment donné pour mieux distinguer ses missions régaliennes de ses missions de gestionnaire d'infrastructure et d'exploitant de service de transport.

Il n'y a aucune référence dans le texte à la notion de filialisation. En revanche, d'autres dispositions de ce type sont d'ores et déjà prévues

afin de maintenir une gestion cohérente et homogène des prestations de sûreté et d'accompagner l'ouverture à la concurrence. Cet article prévoit que les exploitants de services de transport intervenant en région Île-de-France pourront bénéficier de prestations de sûreté fournies par le GPSR. De mon côté, je propose une clarification en distinguant réseaux souterrains et réseaux de surface. S'il existe, pour les premiers, une vraie logique à ce que le GPSR puisse exercer sa mission de sûreté, et ce même lorsque plusieurs entreprises de transport ou exploitants d'installations de services et gestionnaires d'infrastructure sont amenés à intervenir sur le réseau ferroviaire, la situation est différente pour les réseaux de surface, bus et trams. Les prestations des sociétés de sécurité privées ou de services internes de sûreté pour des missions de sécurisation dynamique sont totalement adaptées pour les réseaux de surface, pour un coût d'ailleurs compétitif. Il n'y aurait donc aucune raison de privilégier le GPSR par rapport à d'autres opérateurs de sécurité. Cet amendement a simplement pour objet d'apporter cette précision, tout en laissant la possibilité aux exploitants de recourir au GPSR si le besoin s'en fait sentir dans certains contextes particuliers et selon les enjeux de sûreté auxquels ils sont confrontés. Les trois visant au renforcement de la sécurité des mobilités, qui passe également par une meilleure administration de la lutte contre la fraude. L'application littérale et stricte de l'article L. 2241-1 du code des transports ne permet pas aux agents assermentés de l'exploitant du service de transport d'exercer leurs missions de contrôle des titres et de constatation des infractions aux règles du règlement d'exploitation dans les entreprises qui assurent l'exécution de services en sous-traitance ou non et qui n'ont pas elles-mêmes d'agents assermentés.

assermentés, missionnés par l'exploitant du service de transport. Cette disposition permettrait aux entreprises de transport public de voyageurs de missionner des salariés d'autres entreprises pour procéder au contrôle des titres, salariés qui seraient soumis

Je ne souhaite pas revenir sur ce dispositif, qui garantit un continuum de sûreté dans l'espace et une continuité du niveau de sûreté dans le temps. L'expérience du GPSR, avec les prérogatives dont disposent ses agents, est précieuse à cet égard.

du code des transports conduit à des interprétations trop strictes. Ces amendements offrent de nouvelles solutions aux exploitants de services de transport dans le cadre de la lutte contre la fraude. La commission y est donc

de surface en Île-de-France ne sont pas confrontés aux mêmes risques et n'ont pas les mêmes besoins en termes de services effectuant des missions de sûreté. D'ailleurs, l'article 33 entend répondre à cette préoccupation en permettant l'intervention des agents du GPSR à la demande pour les zones ou les réseaux pour les zones ou les réseaux où leur présence est pertinente. En outre, le code des transports et celui de la sécurité intérieure donnent déjà une grande souplesse aux exploitants de services de transport dans le choix des services et des acteurs. La question du lien entre agents assermentés et exploitants de services de transport est l'objet d'autres amendements, notamment les amendements identiques

Quelque part, on a le sentiment que le texte donne une espèce de priorité ou, en tout cas, accorde davantage de latitude au GPSR pour assurer la sécurité sur l'ensemble des réseaux de transport dépendant d'Île-de-France Mobilités. Je ne reviendrai pas sur le passé : la sécurité dans les transports en Île-de-France était un problème permanent jusqu'à la création de la police régionale des transports et le renforcement des services de la RATP- vous y avez d'ailleurs

? Le I de l'amendement est satisfait par le travail fait en commission pour soumettre la tarification des prestations du GPSR à l'avis conforme de l'Arafer, comme c'est le cas pour la SUGE. Le II Le II prévoit un nouveau schéma de sûreté contraire à la position adoptée en commission. Je rappelle que le GPSR accomplira sa mission de prévention sans préjudice des compétences dévolues à la SUGE de la SNCF sur le Transilien et le RER qu'elle exploite. La coordination entre ces deux services est déjà prévue et organisée, ce qui leur permet d'intervenir sur les sites d'interconnexion des réseaux relevant de la compétence de l'autre service interne de sécurité pour la constatation d'une infraction ou pour l'exercice d'une mission de sûreté après autorisation

Madame la ministre,

: La parole est à M. Alain Fouché. Cette mesure vise à étendre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP l'usage de la force armée en cas de « légitime défense élargie » et de « périple meurtrier

ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes

dans les transports, les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF sont les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir et empêcher immédiatement la réitération d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre.

Le code des transports permet aux agents du GPSR et de la SUGE de porter une arme, après autorisation du préfet. J'attire votre attention sur le fait que le code pénal leur permet déjà de faire usage

accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte » ; en outre, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but visé dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction

Ils ont la possibilité de tirer pour se défendre, dans des cas très spécifiques, au-delà des cas prévus par le code pénal. Aussi, la mesure que vous proposez me paraît aller trop loin : il faut préserver la frontière entre missions de prévention et de sûreté, d'une part, et missions de sécurité, d'autre part.

de la SUGE et du GPSR d'intervenir dans le cadre du « périple meurtrier », ce qui ne relève ni de leurs missions ni de leurs compétences. J'attire votre attention sur le fait qu'une évolution de ce type serait source de risques pour le public et les différentes forces de sécurité,

Madame la ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu'à une heure, afin de poursuivre plus avant l'examen de ce texte. Il n'y a pas d'observation ? ... Il en est ainsi décidé.

Le pouvoir de police générale des maires ne peut pas être transféré aux EPCI. Vous le savez, seuls les pouvoirs de police spéciale peuvent faire l'objet d'un transfert au président d'un EPCI lorsqu'ils se rattachent à l'exercice d'une compétence. C'est par exemple le cas du pouvoir de police de la circulation, qui est un pouvoir de police spéciale, et qui est automatiquement transféré aux EPCI qui sont compétents en matière de voirie. Cet amendement, qui prévoit un transfert du pouvoir de police générale s'agissant des lignes de transport public soulève donc des difficultés juridiques importantes. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Je sais combien l'émotion vécue dans les Pyrénées-Orientales a été partagée par la France entière. Nous sommes toutes et tous convaincus qu'un tel drame ne doit plus jamais se reproduire dans notre pays. J'ai d'ailleurs ressenti un sincère intérêt de la Haute Assemblée sur cette question quand j'ai proposé d'intégrer ma proposition de loi au sein de ce texte de loi d'orientation des mobilités, pour lui donner plus de force et d'efficacité. J'espère de tout coeur que, par nos votes, nous dirons unanimement : « Plus jamais ça ! ». Adoptées à l'entière majorité par notre groupe ainsi qu'au sein de la commission, trois mesures visent à mettre un terme à ces accidents mortels mortels : prévoir que les données sur les passages à niveau soient publiées pour permettre aux fournisseurs de services d'information sur la circulation de s'en saisir et de signaler les passages à niveau aux usagers de la route équiper les véhicules de transport de personnes d'un dispositif d'information sur la localisation des passages à niveau ; réaliser un diagnostic public de sécurité routière des passages à niveau, par l'intermédiaire des gestionnaires de voirie et d'infrastructure ferroviaire. Nous pourrions aller plus loin avec d'autres pistes de progrès : installer des dispositifs de télésurveillance en guise de prévention, de contrôle et de dissuasion ; rehausser les feux à l'approche des passages à niveau privilégier des LED plus visibles ; poser des capteurs de contrôle de fermeture de barrières sur les moteurs ; installer des barrières complètes anti-franchissements ; imposer, dans le code de la route, une obligation de s'arrêter et sensibiliser davantage les auto-écoles. Bien entendu, tout nouveau dispositif de sécurité a forcément un coût, mais que pèse-t-il quand il s'agit de la vie de nos enfants, de nos familles ? De l'avis des experts, ces préconisations pourront être mises en oeuvre sans coût excessif par de nombreux transports déjà équipés en GPS. Devant Fabien Bourgeonnier, le papa du petit Loïc, présent dans notre assemblée ce soir, et au nom de toutes les victimes et de leur famille, c'est donc avec votre coeur, mais aussi et surtout avec votre raison, que je vous appelle, mes chers collègues, à soutenir ces propositions d'une seule et même voix. Je mets aux voix

à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois, une série de mesures destinées à simplifier et à adapter le droit applicable au transport par câbles, notamment les téléphériques et les funiculaires. À l'heure actuelle, les règles régissant la sécurité des installations à câbles sont partagées entre le code du tourisme, s'agissant des installations répondant à la définition d'une remontée mécanique située en zone de montagne, et le code des transports, pour les installations implantées hors zone de montagne. Le règlement européen 2016/424 impose aux États des règles de conception, de construction et de mise en service des nouvelles installations à câbles. à câbles. Il leur impose également d'ouvrir à la concurrence les sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles. Alors que le Gouvernement justifie le recours aux ordonnances par le périmètre limité des remontées mécaniques, la réalité est beaucoup plus large. De nombreux projets de téléphériques se développent en milieu urbain, comme en Isère, à Toulouse ou même en Île-de-France. Le champ du règlement peut s'interpréter comme s'étendant aux installations privées et à celles qui sont situées dans des établissements recevant du public, tels les parcs de loisirs. Dès lors, les procédures d'autorisation, de construction, de modification et de mise en service d'installations à câbles doivent faire l'objet d'une loi en bonne et due forme. La Il est défendu. Quel est l'avis de la commission ? L'objet de l'article 34 est de traiter le cas intermédiaire des installations à câbles situées pour partie en zone de montagne et pour partie en zone urbaine : douze projets de ce type sont à l'étude actuellement-

Les remontées mécaniques de montagne sont prises en compte dans le code du tourisme pour ces équipements qualifiés de « touristiques ». L'ajout d'un cas spécifique aux installations à câbles n'est donc pas utile par rapport à l'objectif visé par les auteurs de l'amendement, car le droit positif prend déjà suffisamment en compte la problématique du bruit causé par les installations à câbles, sans qu'il soit besoin de le modifier. Cet amendement étant satisfait,

Toutefois, la technologie visée n'est pas suffisamment mature pour procéder à une évolution de la réglementation, notamment s'agissant des servitudes d'utilité publique. L'avis est donc défavorable. l'avis du Gouvernement ? Je suis tout à fait favorable au développement de solutions innovantes, mais le principe retenu pour les nouvelles technologies en matière de mobilités est de créer le cadre réglementaire

Ceux-ci sont amenés, quel que soit leur poste de travail, à emprunter ponctuellement ou régulièrement ces remontées mécaniques pour les besoins de leur employeur. À cet effet d'ailleurs, la carte de libre circulation permet de s'assurer du trajet suivi par le salarié et de pouvoir, si besoin, rapidement le localiser pour des raisons de sécurité. Il est impératif, à l'égard des clients empruntant les remontées mécaniques pour leur loisir, que les salariés des exploitants de domaines skiables utilisent les mêmes voies d'accès et, par conséquent, soient munis d'une telle carte. En outre, l'irrégularité de leurs plannings impose aux salariés de bénéficier d'une carte unique de libre circulation, puisque la souplesse d'organisation inhérente à l'exploitation de remontées mécaniques exige qu'un salarié puisse être mobilisé au pied levé pour assurer le remplacement d'un autre salarié sur un poste différent du sien. Or, depuis un récent renforcement administratif, les laissez-passer d'accès aux remontées mécaniques délivrés aux salariés des domaines skiables sont soumis à une taxation par l'Urssaf au titre d'un avantage en nature, pour les charges tant patronales que salariales. En effet, l'Urssaf considère que, même en l'absence d'utilisation d'un forfait ou laissez-passer par le salarié durant ses jours de repos, les deux septièmes du prix du forfait de ski l'usager doivent être imputés comme avantage en nature, alors même que les grilles tarifaires prévoient l'accès gratuit, inclus dans le forfait saison, pour les jours de ski au-delà de vingt-cinq jours. L'avantage consenti est donc nul. Aussi, cet amendement prévoit de supprimer la taxation, réalisée par l'Urssaf, des forfaits de ski utilisés par les salariés des domaines skiables.

du moment où cette carte de libre circulation est également utilisable à titre privé pendant le temps de repos, elle constitue de fait un avantage en nature qui fait partie de la rémunération du salarié. Dès lors, il est normal que cet avantage soit soumis à cotisation, car il ne me semble pas

du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux organise la mise en place de périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture. Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet de retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret. » Cette rédaction qu'aucun dispositif réglementaire ne vient préciser nécessite par conséquent, pour toute réduction de périmètre de PAEN, que la modification soit initiée par le département, qu'elle reçoive l'accord des communes intéressées et qu'elle soit approuvée par décret. La présence d'un PAEN est donc susceptible de fragiliser la création d'infrastructures de transport déclarées d'utilité publique, puisqu'il suffit d'une opposition du département ou de l'une des communes intéressées pour interdire la modification nécessaire à la construction de l'infrastructure. Il convient donc de mettre Il convient donc de mettre en place des outils permettant une telle modification, sur l'initiative de l'État, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics. Le présent amendement vise à permettre de procéder à une modification d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le cadre de la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure linéaire et d'autoriser la poursuite d'un projet sur un secteur qui aurait été classé périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains malgré l'existence préalable d'une réservation foncière préexistante. Cette possibilité est limitée aux seuls projets d'infrastructures de transport de l'État, d'un de ses établissements publics, d'une collectivité territoriale

les collectivités adopteraient des plans de protection dont on pourrait s'exonérer, au gré des décisions d'aménagement de l'État. J'ajoute qu'une telle façon de faire serait même contre-productive, car ces projets d'ampleur ne seront acceptés, sur le territoire, que si un dialogue entre l'État et les collectivités permet de faire émerger un consensus local ; en voulant passer ainsi en force, on risquerait bien plus de freiner les projets. Je rappelle, enfin, que, lors de l'examen de la loi Élan, le Sénat avait fermement défendu la compétence des collectivités en matière d'urbanisme et d'aménagement, contre l'imposition par l'État de projets non concertés. Notre commission est sur la même ligne. C'est pourquoi elle a émis un avis défavorable affirmé

Je voudrais d'abord souligner l'importance des périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, qui peuvent être soumis à des pressions importantes. Ils doivent donc faire l'objet de

n'est pas plus protectrice des préoccupations des communes que ne le serait la procédure qui est proposée par cet amendement. amendement. Cette procédure donne bien toutes les garanties, avec une évolution des périmètres qui est réalisée dans un cadre concerté, itératif et progressif de l'élaboration du projet. Le dispositif proposé permet,, et si certains blocages persistent, de faire évoluer un tel périmètre par le biais d'une DUP. Il prévoit aussi que le dossier indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l'effet du projet d'infrastructure. Il prévoit enfin que ces éléments soient intégrés au dossier d'enquête publique. La procédure est donc tout aussi respectueuse des prérogatives des collectivités et peut se révéler plus efficace pour permettre la prise en compte d'infrastructures de l'État ou d'autres gestionnaires de voiries. C'est pourquoi le

J'aimerais appuyer l'intervention de mon collègue, en rappelant que l'ensemble des départements des Alpes du Nord est favorable à ce trajet également pour les accès au tunnel du Lyon-Turin. est à Mme la ministre. Le Gouvernement est bien sûr mobilisé pour assurer la compétitivité du port de Marseille, notamment ses débouchés au nord de l'Europe, y compris au nord de Lyon.

performants entre Marseille, le nord de la France et de l'Europe, il est aussi important de bien utiliser la voie fluviale. Aujourd'hui, la desserte fluviale ne joue pas tout son rôle, alors qu'il existe un axe

pour permettre à Marseille d'étendre son vers le nord de la France et de l'Europe.

Selon cet article, la convention pourra prévoir de moduler à la baisse une partie du montant de la redevance en fonction du trafic ou de la performance environnementale de la chaîne de transport. Nous souhaitons rendre obligatoire le fait pour la convention de prévoir que le montant de la redevance comportera une part dégressive en fonction du niveau du trafic ou de la performance environnementale. ainsi d'agir efficacement sur les pratiques pour favoriser le report modal vers des modes de transports écologiquement plus vertueux, comme le ferroviaire ou le fluvial. Quel est l'avis de la commission ? C'est C'est un sujet que nous avons vu en commission : le 1° de votre amendement ne laisse aucune souplesse aux parties. Il induirait même un risque de requalification de la convention de terminal en contrat de concession. Le trafic ou la

La croissance des trafics dans les ports maritimes conduit à une augmentation mécanique des acheminements routiers sur des infrastructures déjà saturées, que l'activité ferroviaire et fluviale est orientée à la baisse. La poursuite de cette tendance est susceptible d'entraîner de graves dysfonctionnements dans les ports français. Parallèlement, les infrastructures ferroviaires et fluviales sont largement sous-utilisées. Cette situation affaiblit la position concurrentielle des ports français. Aussi, afin de favoriser et d'engager le report modal vers le transport ferroviaire et le transport fluvial, il convient de réguler les pratiques. Cet amendement vise à aller au-delà de la simple possibilité de prévoir, dans les conventions de terminal, une part dégressive du montant de la redevance en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport. Il tend à prévoir l'obligation d'introduire de telles clauses financières liées à des critères environnementaux. En outre, il vise à supprimer la modulation de la redevance en fonction du trafic, pour ne garder que la modulation en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport. est à Mme Martine Filleul. Cet amendement vise à supprimer la modulation de la redevance en fonction du volume de trafic, pour ne garder que la modulation en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport, la première mesure pouvant être en contradiction avec la seconde, et réciproquement. Il s'agit ainsi de n'encourager que les pratiques vertueuses et respectueuses de l'environnement.

contrat. Mais comment prendre en compte les critères économiques d'évaluation des biens sans exclure pour autant la prise en compte d'autres critères ? En vertu de la pratique courante dans les conventions de terminal, les biens réalisés par l'entrepreneur de manutention sont repris en fin de contrat leur valeur de marché. Il est d'autant plus justifié que l'indemnisation versée à l'opérateur lors du transfert des biens dans le patrimoine du grand port maritime soit fondée sur des conditions, notamment économiques, déterminées d'un commun accord entre les parties : c'est le seul moyen de rassurer les banques prêteuses, dont les financements sont indispensables pour investir à long terme. Sur ce sujet, j'attends une réponse de votre part. Quant au présent amendement, il a pour objet d'encadrer plus strictement le recours de la concession par les grands ports maritimes. L'objectif est de préserver le recours à la convention de terminal.

être utile, et elle serait conforme au droit en vigueur, notamment au considérant 15 de la directive 2014/23 sur les concessions. En revanche, en exigeant de justifier de la nature et de l'étendue de ce besoin, on restreindrait la faculté, pour le port, de recourir à la procédure qu'il estime la plus appropriée.

manutention. Les coûts supportés par les opérateurs fluviaux pèsent de façon croissante sur leur compte d'exploitation. Or l'opérateur fluvial ne maîtrise pas l'opération logistique de bout en bout. Il n'a le choix ni du terminal ni de l'opérateur de manutention. S'agissant du transport routier et ferroviaire, l'ensemble des coûts de manutention portuaire est facturé au donneur d'ordre. Cette différence de traitement entre les opérateurs n'existe pas dans les ports concurrents des pays du nord de l'Europe, dans lesquels la part du transport fluvial est plus importante que celle des grands ports maritimes français. Le transport fluvial en France s'en trouve non compétitif et discriminé par rapport au transport au transport routier ou ferroviaire. Pour remédier à cette anomalie, nous proposons, par cet amendement, de généraliser une solution retenue pour le grand port maritime de Dunkerque : inclure les coûts de manutention fluviale dans les charges et les facturer au donneur d'ordre.

a pu être mis en place sur un volume assez restreint de marchandises. Toutefois, la précision que vous proposez est contraire à l'esprit de la réforme portuaire de 2008 et au texte adopté en commission, qui prévoit une dérogation à l'ordonnance Concessions sur les tarifs à la charge des usagers. L'alinéa 6 de l'article 35 vise précisément à éviter un contrôle tarifaire de l'activité du manutentionnaire

Cet amendement tend à associer la commission des investissements aux orientations du grand port maritime en matière de concessions et de conventions de terminal. On approfondirait ainsi le dialogue entre les acteurs de la place portuaire autour du développement économique, sans alourdir la procédure de passation des contrats pour les grands ports maritimes et en évitant de potentiels conflits d'intérêts pour les membres de la commission des investissements. Il s'agit évidemment de faire en sorte que l'ensemble des opérateurs des grands ports français, non seulement se parlent, mais essayent de travailler mieux ensemble.

ministre. Cet amendement a pour objet d'assouplir les règles de connaissance du français par les capitaines et suppléants, afin d'encourager le passage sous pavillon français des navires.

les armateurs qui souhaiteraient placer des navires sous pavillon français doivent pouvoir disposer d'une période transitoire pour recruter et former des marins francophones.

Cette mesure a fait l'objet de discussions avec les professionnels du transport maritime. Nous l'avons d'ailleurs évoquée récemment au sein du groupe d'études Mer et littoral, que préside notre collègue Michel Vaspart, avec les représentants

Au regard des bénéfices économiques, environnementaux et sociaux que représente le canal Seine-Nord, nous nous attendions à ce que l'État rôle structurant dans le financement global de cette infrastructure. Or le temps passe et, à ce jour, aucune maquette budgétaire stabilisée et complète n'a été finalisée. Il est pourtant urgent de la présenter à l'Union européenne, qui est prête à financer 50 % des travaux, et aux collectivités territoriales concernées, qui ont démontré leur attachement à ce projet.

et non prélever une nouvelle taxe sur les habitants de la région. Il est urgent, maintenant, que le Gouvernement s'implique. Les députés et les sénateurs concernés demandent également la nomination d'un délégué interministériel pour

comprenant notamment des élus, des représentants de la société civile, ainsi que des représentants des professionnels concernés par l'exploitation et l'utilisation de l'infrastructure. Quel

I, lequel prévoit la réalisation du canal Seine-Nord. Je peux vous assurer que le travail est en cours : ne doutez pas que le ministre de l'action et des comptes publics est particulièrement mobilisé pour trouver une solution.

relative à la société du canal Seine-Nord Europe prévoient d'ores et déjà la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil de surveillance de l'établissement et la création d'un comité stratégique auprès de celui-ci. L'habilitation proposée à l'article 36 ne conduira à revenir ni sur cet aspect de la composition du conseil de surveillance ni sur la composition du comité stratégique : il s'agit uniquement de modifier la répartition des représentants des collectivités territoriales et des représentants de l'État au sein du conseil de surveillance, de façon à conférer la majorité des voix aux collectivités territoriales.

dire, nous parlons depuis de nombreuses années déjà. Nous notons quand même avec satisfaction que, au fil des années, l'intervention de l'Europe a été

la participation de l'Europe s'élève à 50 % de l'ensemble du projet. Les collectivités territoriales se sont fortement mobilisées, et avec une certaine

toutes tendances politiques confondues, les clefs de répartition qui nous ont permis d'être à ce rendez-vous. Oui ! De plus, M. Bascher vient de faire état du fonctionnement de la société de projet, de l'implication du président Xavier Bertrand et de l'ensemble des élus qui y siègent, notamment

Martine Filleul démontre s'il en était encore besoin que, de manière transpartisane, l'ensemble des acteurs de ce dossier sont fortement impliqués, et depuis longtemps.

Tel est bien le rôle de ces schémas : fixer des orientations générales d'aménagement régional. La mesure proposée permettrait de renforcer la cohérence, à l'échelle régionale, des politiques publiques menées par les collectivités territoriales en la